Monsieur le président, La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 15 avril 2020 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de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

doit nous permettre de faire face aux exigences économiques nouvelles liées à la crise du coronavirus. Je voudrais d'abord rappeler

avec d'ailleurs une inquiétude particulière, à présent, pour les pays en voie de développement et les pays africains ; une récession qui se chiffre,

risque pour la transition énergétique, car pour réussir celle-ci, encore faut-il que les prix des énergies fossiles soient à un niveau raisonnable et que nous puissions financer les énergies renouvelables

Face à cette situation économique sans équivalent dans l'histoire contemporaine, nous avons voulu, avec le Président de la République et le Premier ministre, prendre immédiatement la mesure de la crise. Nous avons immédiatement dit la vérité aux Français : cette crise économique est l'une des plus graves que nous ayons connues depuis la grande récession de 1929. Les fondamentaux ne sont pas les mêmes, les logiques non plus, les réactions des États non plus, mais la profondeur de la récession est comparable à ce que nous avons connu en 1929. Nous avons toujours tenu ce langage de vérité, depuis le premier jour de la crise économique : nous n'en avons jamais dissimulé ni la gravité ni les conséquences. Nous avons aussi voulu apporter une réponse rapide, forte et immédiate. Nous avons fait un choix très simple, que nous revendiquons devant la représentation nationale, devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs de la dette plutôt que des faillites ; de la dette plutôt que la disparition de décennies entières d'efforts économiques des salariés, des ouvriers, des employés, des ingénieurs et des entrepreneurs français. Ce choix, je le revendique

Nous vous proposons donc aujourd'hui, par le biais de ce projet de loi de finances rectificative, d'une part de recharger le dispositif existant, parce qu'il coûte cher, et d'autre part de l'améliorer.

Enfin, concernant les entreprises stratégiques, vous nous avez fait observer à juste titre que le compte d'affectation spéciale (CAS) destiné à les soutenir était insuffisamment doté pour apporter du capital aux entreprises qui en auraient besoin ; nous avons donc décidé d'augmenter de 20 milliards d'euros

Mais l'économie française devra fonctionner autrement dans les mois qui viennent. Il faudra commencer par redémarrer, par reprendre l'activité, reprendre le chemin du travail. C'est la demande qui m'a été faite par le Premier ministre et le Président de la République : examiner comment nous pouvons faire redémarrer l'économie française dans des conditions de sécurité sanitaire totale ce dernier mot. Je ferai donc des propositions au Premier ministre et au Président de la République dans les heures qui viennent, en essayant d'offrir aux

aux secteurs de l'alimentation, de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution, qui ont tourné, contre vents et marées, malgré les difficultés et les risques sanitaires ; les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, les agents de caisse, les metteurs en rayon, les transporteurs, tous étaient là, fidèles au poste, pour garantir la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et une vie à peu près normale.

et je pense que n'importe quel Français, dans son lieu de travail, dans les lieux de culture, dans n'importe quel lieu d'activité, dirait exactement la même chose. Mais il se trouve que, pour des raisons de sécurité sanitaire, nous devons vivre avec de la distance. Or dans les lieux de convivialité que sont les restaurants, les bars, ou les cafés, le défi est beaucoup plus considérable que dans n'importe quel autre lieu d'activité professionnelle. Il faudra donc se donner un peu plus de temps

dans des conditions de sécurité sanitaire totale, de manière à ce que leurs clients soient rassurés et à ce que leur activité puisse se poursuivre. Nous prendrons donc le temps nécessaire pour garantir la réouverture dans les meilleures conditions possible de tous les restaurants, de tous les bars et de tous les cafés français. La troisième et dernière étape, après la réponse immédiate et la reprise progressive du travail, sera la relance de notre activité économique. Il faut y penser dès maintenant

La première ligne directrice de cette relance est l'investissement. Ce qui va manquer à l'économie française, aux entreprises françaises, aux technologies françaises, à notre industrie, c'est de l'investissement. Aujourd'hui, il est à zéro,

Il faut nous assurer que les Français retrouvent le goût de la consommation et que la demande reparte ; sinon, notre économie aura du mal à redémarrer rapidement.

Aujourd'hui, le Gouvernement table sur un recul de plus de 8 % du PIB ; c'est sans doute beaucoup plus réaliste et cela constitue, Gérald Darmanin vient de le dire, la pire performance depuis l'après-guerre.

héritage budgétaire ne paraît pas de nature à remettre en cause la soutenabilité de la dette française, à condition que, bien entendu, une fois cette crise passée, nous soyons capables de redresser les comptes publics. Le budget que vous nous présentez, messieurs les ministres, est, je le dis

Les chiffres, nous en convenons tous, sont vertigineux, mais je crois que la situation l'exige. Logiquement, c'est la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » qui connaît l'augmentation la plus

nous trompons pas de tempo, nous aurons des propositions à faire sur la relance, mais, aujourd'hui, nous sommes dans le sauvetage et nous souhaitons y contribuer par nos amendements. La parole chers collègues, nous voici en séance pour examiner un deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2020, exactement un mois après l'examen du précédent. Cet exercice était déjà annoncé lors de nos débats du mois de mars ; nous le pressentions, cela s'est confirmé. Très vite, les chiffres présentés dans le premier PLFR- une croissance en baisse de 1 %, un déficit de 3,9 % du PIB, une dette publique en légère hausse -se sont révélés en décalage par rapport à l'ampleur de la crise que nous traversons. Les pertes de recettes fiscales étaient largement sous-estimées, de même que le coût budgétaire du dispositif de chômage partiel. Dans le présent texte, la chute du PIB est désormais estimée à 8 %, le déficit public serait porté à 9 % du PIB et la dette consolidée à 115 % du PIB. Même s'il s'agit d'un constat sévère et d'une dégradation historique de nos finances publiques, même si, à cette heure, toutes les estimations doivent encore être considérées avec prudence, cet exercice de sincérité des comptes était nécessaire ; il est donc le bienvenu.

De même, la crise affecte l'ensemble des politiques publiques et son effet, à la hausse, mais parfois aussi à la baisse, avec un décalage de certaines dépenses- je pense par exemple aux investissements qui ne peuvent être engagés -, devrait être mesuré. Il ne suffit pas d'affirmer que les ouvertures de crédits budgétaires, annoncées par tel ou tel membre du Gouvernement, seront financées par des économies de constatation ; ces données devront être présentées au Parlement. Il n'est pas envisageable ni raisonnable, du point de vue du pilotage de l'action publique, d'attendre le schéma de fin de gestion pour faire les comptes de chaque mission budgétaire. Ce projet de loi de finances rectificative permet également de répondre aux observations sur l'insuffisance du premier plan d'urgence, que beaucoup d'entre nous avaient pointée.

Les mesures pour le personnel soignant et le soutien aux ménages modestes étaient également attendues. Pour autant, chacun sait que le deuxième PLFR n'est encore qu'une étape ; un troisième projet est d'ores et déjà en préparation, nous dit-on. Il sera celui des arbitrages politiques. Quel sera le plan de relance ? Quels secteurs seront prioritaires ? Surtout, après avoir constaté la sévérité de la crise et de son impact sur nos finances publiques, avec une hausse de la dette publique de près de 20 points de PIB, comment financer cette relance ? Malgré l'accord survenu à Bruxelles, il n'existe pas encore de plan européen de relance ; jusqu'où pourra-t-on aller, à l'échelon national, sans un fort soutien européen ? Pour ce qui concerne la part de financement national,

Je souhaiterais également que le prochain PLFR prenne en compte la situation des collectivités territoriales, dont les recettes sont très fortement touchées, qu'il s'agisse des redevances

du fonds de solidarité, consistera à mettre en place des dispositifs spécifiques à certains secteurs : le tourisme, la culture, l'événementiel, l'hôtellerie et la restauration ». Nous espérons pouvoir examiner ces mesures rapidement, tant ces secteurs sont durement frappés. Au-delà de ces branches, nous souhaitons une prise en compte de la situation des entreprises, quel que soit le secteur, dont les charges fixes non modulables sont élevées. À l'heure où nous débattons de ce texte, beaucoup d'incertitudes demeurent, et non des moindres, sur les conséquences de la crise sanitaire qui a conduit à mettre notre pays pratiquement à l'arrêt. Le Gouvernement nous demande de lui faire confiance, tant pour les initiatives qui devront être prises pour le redémarrage de l'économie que pour les mesures de sauvetage qu'il devra mettre en oeuvre, en ouvrant 20 milliards d'euros supplémentaires pour permettre des recapitalisations, sans connaître les entreprises concernées ni le calendrier de mise en oeuvre.

Tout le monde, du moins en France et en Europe- peut-être à une exception près, du côté de la Biélorussie -, s'accordera sur cet impératif sanitaire. Toutefois, notre pays doit aussi être vigilant à l'égard de son économie et de son fonctionnement social, qui contribuent également à la santé de nos concitoyens. pour les semaines, les mois et peut-être les années à venir, est aussi incertain que le scénario sanitaire. Le premier dépend en partie du second, mais pas seulement, et les incertitudes persistantes ne doivent pas brider notre capacité d'action et d'initiative. Dans l'urgence, nous avons adopté conforme, au mois de mars, un premier PLFR, qui avait un caractère certes incomplet, mais qui avait le mérite de mettre en place les principaux outils d'intervention permettant d'éviter un effondrement de l'économie, la disparition de nombreuses entreprises et une explosion du chômage. Je pense en particulier au dispositif immédiatement mis en place et très vite opérationnel du chômage partiel. J'aurai toutefois une question à ce sujet : lorsque l'on parle de près de 10 millions

Dans ma question au Gouvernement du 1 avril dernier, j'estimais, messieurs les ministres, que le dispositif adopté méritait d'être amplifié, complété et parfois précisé, et j'appelais à la mise en place d'un fonds de solidarité beaucoup plus ambitieux. Les réponses que nous trouvons dans le PLFR 2 répondent assez positivement à ces remarques.

ont fait l'objet d'assouplissements et que les mesures sectorielles visant les professions se trouvant dans l'incapacité de reprendre prochainement leur activité ne semblent pas- c'est normal -avoir été totalement intégrées à cette montée en puissance. Il convient aussi de se féliciter de dispositions complémentaires importantes, comme la dotation supplémentaire de 925 millions d'euros au Fonds de développement économique et social, pour l'octroi de prêts à des entreprises fragiles ou en difficulté et dont le redressement nécessite une restructuration. Avec un engagement financier d'une autre dimension, la mission « Participation financière de l'État » est dotée de 20 milliards d'euros de crédits, pour renforcer les fonds propres d'entreprises stratégiques. C'est une mesure indispensable.

Tout en respectant les mesures de protection sanitaire, notre économie aurait sans doute pu maintenir un niveau d'activité plus élevé que celui que nous avons connu au cours des dernières semaines ; on ne va pas refaire l'histoire, mais un certain nombre d'entreprises, y compris publiques, comme La Poste, ont été très réactives pour mettre le pied sur le frein Le redémarrage risque d'être hétérogène, suivant la nature des activités, et sans doute un peu chaotique, à la veille d'un été qui suscite bien des interrogations.

même avec un regain dynamique d'activité, je ne vois pas comment ces entreprises pourraient être en mesure, en juillet ou en septembre, de faire face à un double montant d'échéances. Ce dispositif existe ; autant s'appuyer dessus. Nous devrons aussi, au cours des prochaines semaines, anticiper, peut-être avec des mesures complémentaires, la reprise, sans doute très progressive, de secteurs d'activité touchant au tourisme, aux loisirs, à la restauration, à la culture et au sport. Je souhaite que nous puissions aborder la renaissance de ces secteurs lors de notre prochaine réunion, pour examiner un PLFR 3, ce qui serait bien évidemment un excellent signe.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, sans surprise, je vais voter les crédits du deuxième PLFR. Ne vous y trompez pas, messieurs les ministres, il s'agit de faire en sorte que vous disposiez des moyens financiers pour répondre aux trois défis que cette situation exceptionnelle nous impose : le défi sanitaire, le défi économique et le défi sociétal. Le défi sanitaire est loin d'être gagné et si, dans cette période, il n'est pas question d'entrer en polémique, il faudra bien faire un jour le bilan de vos décisions. Je pense notamment aux tests. Tous les pays qui ont maîtrisé au mieux leur situation ont eu une politique massive de tests. En France, il semblerait que l'on s'interroge encore sur lequel choisir Tous les retards de décision auront un coût humain et financier, et le Gouvernement en est responsable puisque nous lui en donnons les moyens. En matière économique, là aussi, nous sommes d'accord pour que vous puissiez disposer des marges de manoeuvre nécessaires, mais nous devrons comparer l'utilisation de ces moyens avec la pratique de nos voisins. Force est de constater, par exemple, que nous consacrerons trois fois plus de moyens au chômage partiel que l'Allemagne,

On voit bien qu'une chose est de disposer de moyens financiers, une autre est la mise en oeuvre des stratégies. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de vous donner les moyens d'une politique forte. Vous serez responsables de la qualité de sa mise en oeuvre. Les Français ont de plus en plus de mal à se tenir confinés. L'espoir d'un rebond fort peut les aider à tenir, mais ne nous y trompons pas : si la problématique santé est prioritaire, les dégâts sociétaux consécutifs à une économie chancelante pourraient être considérables. Les Français sont nombreux à s'interroger sur les effets de la valse des milliards. Ceux qui pensent que cela n'aura pas de conséquence se trompent. Demain plus que jamais, nous aurons besoin de citoyens forts, entreprenants, responsables et n'attendant pas tout de l'État.

l'examen d'un projet de loi de finances rectificative ne permet évidemment pas d'embrasser tous les aspects d'une loi de finances initiale. Nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire, sociale et économique. Cependant, les mesures qui s'inscrivent dans ce PLFR devraient déjà, selon nous, donner des signes clairs quant aux politiques qui seront menées demain. Les choix du moment devraient engager fortement l'avenir de notre société. Le Gouvernement a décrété d'emblée que notre fiscalité ne serait pas modifiée. Cette crise sanitaire bouscule la planète entière, notre continent européen, et percute de plein fouet la société française, qui souffre de fortes inégalités depuis trop longtemps. L'Insee montrait qu'en 2018 la pauvreté avait augmenté de 0,6 % dans notre pays ; personne ne niera que le confinement est beaucoup plus difficilement supportable quand on est confronté au mal-logement ou à l'absence de moyens numériques pour assurer la continuité éducative des enfants. Cette crise met aussi en évidence la nécessité de services publics forts, celui de la santé d'abord, de l'éducation aussi, ou encore des collectivités locales. Les discours du Gouvernement, dans la période, tranchent singulièrement avec certains propos tenus au début de ce quinquennat.

M. le ministre Bruno Le Maire, ici présent, lui emboîtait le pas quelques jours plus tard avec ces paroles : « Depuis trente ans, la France est droguée aux dépenses publiques. Oui, il faut les réduire : c'est une question de souveraineté nationale. Enfin, et j'arrêterai là mon inventaire, la fameuse formule du président Macron, en juin 2018 : « On met un pognon de dingue dans les minima sociaux ». Ces propos pourraient-ils encore être tenus aujourd'hui, en pleine crise sanitaire où la dépense publique devient un outil essentiel ? Nous considérons pour notre part que les prochains débats budgétaires se tiendront dans un contexte profondément modifié, où les repères libéraux auront été largement bousculés. Vous faites le choix de financer vos mesures par la dette, et nous avons même entendu un temps très bref un appel à la générosité publique. Or la force d'un État, c'est notamment sa capacité à lever l'impôt. Nous pensons qu'il y a des ressources à solliciter du côté des plus gros patrimoines, des plus hauts revenus, ou encore des dividendes, dont le niveau a battu un record l'an dernier avec 51 milliards d'euros, un chiffre qui fait de la France le meilleur rémunérateur d'actionnaires en Europe. Notre groupe a déposé plusieurs amendements visant à solliciter ces ressources. Les aides aux entreprises ne sauraient se limiter aux plus grands groupes industriels stratégiques ; il faudra veiller à ce que l'ensemble du tissu économique soit demain en mesure de retrouver rapidement sa vitesse de croisière. Il importe également de conditionner ces aides. L'on ne saurait imaginer l'octroi d'argent public à des groupes qui distribueraient des dividendes, pratiqueraient des licenciements ou auraient des liens avec les paradis fiscaux. À la date d'aujourd'hui, on estime que la dette de la France pourrait atteindre 115 % du PIB.

Dans cette crise internationale, on a vu des tabous tomber. La banque centrale britannique a pris la décision, le 9 avril dernier, de financer directement le Trésor afin de l'aider à affronter les ravages sanitaires et économiques provoqués par l'épidémie de Covid-19. C'est bien un pilier de la doxa libérale qui s'effondre, à savoir l'indépendance des banques centrales et l'interdiction qui leur est faite de financer directement les États. La Réserve fédérale aux États-Unis a suivi le même chemin et a déjà engagé des moyens illimités pour soutenir l'économie du pays. Il faudra bien à un moment donné lancer ce débat de fond au niveau européen. Il faudrait, dans les circonstances présentes, redéfinir fondamentalement le rôle de la Banque centrale européenne. Notre pays va donc encore enrichir les marchés financiers et nous ne connaîtrons pas davantage les détenteurs ultimes de nos titres de dette. Avouez que la souveraineté de la France est singulièrement mise en danger ! Les collectivités locales doivent être également particulièrement aidées, pour deux raisons essentielles elles sont d'abord, avec beaucoup d'autres, aujourd'hui en première ligne, prenant les initiatives les plus diverses pour soutenir et accompagner les populations dans cette crise ; ensuite, ces collectivités seront demain des leviers essentiels dans le redémarrage économique de notre pays- rappelons qu'elles représentent encore 73 % de l'investissement public. Elles ne doivent plus à l'avenir être considérées comme des variables d'ajustement à la baisse de la dépense publique. Enfin, les aides aux plus démunis dans ce PLFR ne sont pas à la hauteur des enjeux du moment, comme les efforts pour les personnes bénéficiant des minima sociaux, sans compter les demandeurs d'emploi non indemnisés, ainsi que les étudiants boursiers. Nous nous étonnons également de l'absence, dans ce PLFR, de mesures d'ampleur pour l'éducation nationale. Certes, on y évoque une prime aux enseignants qui ont assuré l'accueil des enfants du personnel soignant, mais la problématique est, selon nous, beaucoup plus globale. L'école, dans ce pays, représente 12 millions d'élèves et 800 000 personnels. Il faudra sans doute, dans un prochain PLFR, prendre des mesures fortes pour aider les élèves en décrochage dans cette période difficile à retrouver le chemin de la réussite, car on connaît l'incidence forte de la sociologie sur la réussite scolaire des élèves. Ainsi donc,

un déficit maintenu à 2,2 % du PIB, une dette stabilisée à 100 %, une croissance à 1,2 % ... Rarement loi de finances initiale aura été rendue caduque aussi rapidement, et dans de telles proportions Le déficit qui plonge à 9 % du PIB, la dette qui s'envole et la récession qui frappe à-8 % : telle est désormais la réalité avec laquelle nous devons composer. La froideur de ces chiffres a de quoi nous glacer le sang. Nous espérons tous que les conséquences sanitaires de la pandémie seront rapidement limitées, et je souhaite ici m'associer à la douleur de tous nos concitoyens pour qui la période du confinement est aussi celle d'un deuil. Grâce à la mobilisation exceptionnelle de nos soignants, de nos chercheurs et de tout le pays, je suis certain que nous vaincrons le virus. Cependant, nous savons désormais que les conséquences économiques de la pandémie grèveront longtemps nos finances publiques. Et pour cause : les moyens nécessaires que nous mobilisons pour sauver nos entreprises donnent le vertige. Alors que nous nous apprêtons à voter un projet de loi de finances rectificative qui entérine une dette à 115 % du PIB et sanctionne une dépense publique au-delà de 60 % du PIB, je tiens à le rappeler : la situation est alarmante. Pourtant, nous devons nous rendre à l'évidence : sans entreprises, pas de reprise. Telle doit être aujourd'hui notre seule préoccupation préserver le tissu de nos entreprises ; aider nos artisans, nos TPE, nos PME, nos ETI et nos grandes entreprises à passer la crise, à tenir bon, à survivre, ni plus ni moins. La santé a commandé hier la stratégie du confinement pour tous les citoyens. Ce n'est pas terminé, mais l'économie commande aujourd'hui la stratégie du soutien pour les entreprises en difficulté. Au vu de la situation actuelle, le plan de sauvetage de 110 milliards d'euros apparaît malheureusement comme une impérieuse nécessité- une impérieuse nécessité, certes, mais nous devons garder à l'esprit que nous n'avons pas cet argent. Le plan que nous votons aujourd'hui sera donc financé par les générations futures. C'est encore ce que nous avons de mieux à faire, car mieux vaut transmettre un actif et un passif, c'est-à-dire un bilan, une entreprise, que pas d'entreprise du tout. Mais les générations qui naîtront dans le monde de demain paieront les décisions que nous allons prendre aujourd'hui. Soyons-en conscients. Le dispositif de chômage partiel s'inscrit dans cette logique. Il s'agit d'une mesure sociale qui s'avère indispensable par la souplesse qu'elle accorde aux entreprises. Elle permet de sauvegarder aujourd'hui les emplois dont nous aurons besoin demain pour relancer l'activité du pays. Le renforcement des deux dispositifs exceptionnels mis en place lors du premier PLFR, le chômage partiel, que je viens d'évoquer, et les prêts garantis par l'État, me semblent aller dans le bon sens : l'État prend à sa charge le financement des conséquences liées à la crise, sans chercher à tout administrer. Le renforcement de ces dispositifs répond aux attentes des acteurs du terrain. Il en va de même pour la dotation du fonds de solidarité. En totalisant l'abondement supplémentaire de l'État, le concours des régions et la participation des assureurs, désormais un peu plus en phase avec la gravité de la situation, le fonds est aujourd'hui doté de plus de 7 milliards d'euros. Ce rehaussement, accompagné d'une révision des critères d'éligibilité, répond aux attentes du terrain, notamment dans les territoires les plus fragiles. Un mot, enfin, sur les futures prises de participation de l'État au capital d'entreprises stratégiques. Je salue cette décision indispensable qui matérialise notre souveraineté économique, et je ne doute pas que ces participations seront aussi temporaires que possible. Je regrette seulement que le Parlement ne puisse pas, à ce stade, participer plus activement à la définition de cette stratégie, même si j'en comprends les raisons. Je rejoins en cela la position du rapporteur général Mes chers collègues, en votant le premier PLFR, nous nous doutions bien qu'il y en aurait un deuxième. Et en abordant le deuxième, on ne peut qu'envisager un troisième

Cette catastrophe sanitaire entraîne dans son sillage une catastrophe économique qui explique que nous nous retrouvions ici pour un second projet de loi de finances rectificative, à peine plus d'un mois après en avoir adopté la première mouture. Dans un contexte exceptionnel où les inconnues sont nombreuses, mesurer l'ampleur des dégâts relève de la gageure. Le groupe Union Centriste a salué, en mars dernier, la réactivité du Gouvernement, dont la réponse a permis tout à la fois de protéger les salariés et de soulager la trésorerie des entreprises en difficulté. Compte tenu du prolongement du confinement, dont le coût hebdomadaire pour l'économie française est chiffré à près de 20 milliards d'euros par l'Insee, la situation d'un grand nombre de nos entreprises, dans un grand nombre de secteurs, s'est aujourd'hui fortement détériorée. Dans le présent « collectif budgétaire », le Gouvernement propose de porter de 45 milliards à 110 milliards d'euros le plan d'urgence économique. Le budget dédié au dispositif de chômage partiel voit ainsi ses crédits quasiment tripler, pour atteindre désormais 24 milliards d'euros. C'est une somme considérable, mais non moins nécessaire. De même, les crédits alloués au fonds de solidarité pour les TPE sont revus très nettement à la hausse, à 7 milliards d'euros. Il faut s'en réjouir. Ce budget rectificatif instaure également un dispositif exceptionnel de soutien aux prêts et aux fonds propres, à hauteur de 20 milliards d'euros, pour les entreprises dites « stratégiques fragilisées par la crise. Il faudra veiller, messieurs les ministres, et nous y veillerons, à ce que l'État n'investisse pas à fonds perdu dans des activités commerciales en subventionnant aveuglément les investisseurs et les créanciers de ces grandes entreprises. Il est en tout cas heureux que l'Assemblée nationale ait subordonné le soutien de l'État, et à travers lui celui des contribuables, au respect d'objectifs environnementaux. Nous approuvons cette mesure et espérons qu'elle prospérera à l'issue de la navette parlementaire. Le Gouvernement a fait le choix opportun de plusieurs mesures complémentaires, à la fois bancaires, budgétaires et fiscales, visant opportunément à sauvegarder l'appareil productif français et il faudra aller plus loin s'agissant de certaines d'entre elles. Nous l'avons dit le mois dernier : le report des échéances sociales et fiscales était nécessaire. Mais il est devenu insuffisant à mesure que s'est prolongé le confinement. Nous avons appris, lors de la présentation de ce PLFR « nouvelle version », que 750 millions d'euros allaient être consacrés à des annulations de charges sociales et fiscales, dans le cadre de plans sectoriels concernant l'hôtellerie, la restauration ou encore l'événementiel. Mes collègues du groupe Union Centriste et moi-même pensons qu'il sera tôt ou tard inévitable de transformer ce report en annulations pures et simples. Nous déposerons en ce sens un amendement, sans limitation sectorielle, mais à la condition que soient satisfaits certains critères rigoureux, notamment celui du chiffre d'affaires. Notre volonté est non seulement de réserver le bénéfice de cette annulation aux entreprises les plus en difficulté, mais aussi d'en limiter le coût pour les finances publiques. Nous approuvons évidemment le versement d'une prime exceptionnelle aux agents publics mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Cette prime est une juste reconnaissance du travail effectué, s'agissant en particulier des personnels hospitaliers. Mais, pour être tout à fait justes, il nous faudrait aussi marquer notre reconnaissance à tous les autres : songeons en effet aux médecins généralistes, infirmières et infirmiers libéraux, salariés de laboratoires d'analyses et de dépistages, et à toutes celles et tous et tous ceux qui, au péril de leur vie, allant même jusqu'à la donner, ont affronté le danger sans réserve ! Ne pourrait-on pas, messieurs les ministres, prévoir un nouveau dispositif ou calibrer les dispositifs existants de façon à rétribuer leur vaillance ? Nous le savons, et le rapporteur général l'a rappelé ce matin en commission des finances : la saison des PLFR ne fait que commencer. À travers cet épisode 2, le solde budgétaire se dégrade déjà, par rapport à la loi de finances initiale, de 92 milliards d'euros, pour s'établir à plus de 185 milliards d'euros. « Une fois qu'on a passé les bornes, il n'y a plus de limites », écrivait Alphonse Allais. Mais que ce soit par le canal budgétaire ou le canal monétaire, par la voie nationale ou la voie européenne, chaque euro injecté devra un jour ou l'autre être remboursé. Notre collègue Nathalie Goulet, rapporteur spécial des crédits de la mission « Engagements financiers de l'État », vous l'expliquerait mieux que moi. Espérons ainsi que nos débats de ce jour permettent d'esquisser le plan d'investissement qu'il nous faudra, sans tarder, collectivement bâtir pour éviter chacun des écueils. Cela dépendra évidemment des perspectives de la sortie de crise. L'hypothèse privilégiée par le Gouvernement d'un retour rapide à la normale, avec une consommation rebondissant dès le second semestre, nous paraît plutôt optimiste. Les exemples récents sont là pour nous montrer que thésauriser est souvent le premier réflexe après les périodes de tumulte. Nous devrons nous méfier de « la relance pour la relance », souvent dispendieuse. L'épargne devra être drainée le plus rapidement et le plus efficacement possible vers le tissu productif. Au-delà du choc sanitaire et économique qu'elle provoque dans le pays tout entier, la pandémie de Covid-19 aura un impact particulièrement lourd sur l'ensemble des collectivités territoriales qui, grâce à la proximité des élus locaux avec les administrés, grâce aussi à leur réactivité et leur agilité, ont démontré le rôle primordial qu'elles savaient jouer en ces circonstances si singulières. Pour que leurs initiatives se poursuivent et produisent tous leurs fruits, il faudra veiller, messieurs les ministres, à leur conférer les outils juridiques et financiers leur permettant d'accompagner au mieux nos campagnes, nos villages et nos villes de province L'examen du texte par l'Assemblée nationale a déjà permis de notables progrès. Parmi ceux-là, nous nous félicitons de l'abaissement du taux de TVA applicable aux gels hydroalcooliques ainsi qu'aux masques de protection, mesure réclamée par notre président Hervé Marseille. Nous espérons que l'examen de ce PLFR par la Haute Assemblée permette, dans un esprit toujours constructif, de préserver la vitalité et les forces de notre pays. Enfin, en votre nom à tous, vous me permettrez d'avoir une pensée pour tous nos malades, qu'ils soient hospitalisés ou isolés dans leur domicile. Personne ne s'adresse jamais à eux Depuis le début de la crise sanitaire, les malades sont devenus des chiffres ou, pire, ont disparu parce que non comptabilisés. Le Sénat n'étant pas une assemblée à chiffres, adressons donc à tous les malades notre soutien et nos espoirs, notre énergie aussi, parce que leur combat vaut largement le nôtre cet après-midi !

Très similaire, car le pays est toujours confiné et nous sommes toujours en train de lutter contre cette maladie qui le paralyse largement. Mais aussi très différent, car ce deuxième texte nous est soumis alors que nous en savons aujourd'hui davantage sur les conséquences économiques possibles de la pandémie. Lors du premier PLFR, notre groupe, par la voix de Thierry Carcenac, avait fait part de ses réserves sur le cadrage macroéconomique présenté par le Gouvernement. Les données présentées dans ce deuxième texte le confirment : 9,1 % de déficit attendu pour 2020, 115 % de dette et 8 % de récession. Nous espérons tous que ces chiffres pourront être revus positivement dans les semaines et les mois qui viennent, en tout cas qu'ils ne s'aggravent pas encore, mais ce scénario semble à ce stade cohérent et pertinent. Se pose dès lors la question, parmi mille autres, de l'impact de la stratégie de déconfinement sur la reprise de l'activité économique. même si je conviens qu'il ne s'agit pas du coeur du sujet, que nous partageons les craintes exprimées par le Haut Conseil des finances publiques : estimer que l'essentiel de l'impact économique concernera le premier semestre de l'année et que le retour à la normale pourrait être rapide et complet nous semble être un pari certes positif, mais risqué quant à l'avenir ... et au niveau de nos finances publiques. Puisque nous abordons la question des chiffres, je voudrais également vous mettre en garde, messieurs les ministres, comme nous l'avons fait dès le premier PLFR, sur le vocabulaire qu'emploie le Gouvernement durant cette crise. Le climat est suffisamment anxiogène pour nos concitoyens pour ne pas ajouter, au-delà des polémiques portant sur la gestion de la pandémie, celles sur les chiffres. Laisser penser que vous injectez 110 milliards d'euros est une manière particulièrement biaisée de présenter les choses. Il y a tout d'abord les 20 milliards d'euros de participations financières de l'État dont on ne sait pas encore s'il s'agit d'une dépense réelle. À ce stade, il s'agit avant tout d'une provision permettant d'agir autant que de besoin pour renforcer nos entreprises. De plus, l'expérience passée montre que ces prises de participation sont, au final, rentables pour l'État. Il y a également 50 milliards d'euros qui relèvent d'avances de trésorerie et pas de dépenses réelles. Il y a également 8 milliards d'euros, au bas mot, qui sont assumés non pas par l'État directement, mais par l'Unédic, même si l'État en assume le portage à ce stade, et 8 milliards d'euros qui sont portés par le budget social et non par le budget général de l'État- je reviendrai plus loin sur ce point. Je vous épargne l'analyse au milliard près, mes chers collègues, mais je crois que tout le monde comprend l'idée générale n'en faisons pas trop avec les chiffres, messieurs les ministres, ou plus exactement adoptons moins d'emphase et plus de sobriété dans le discours sur ce point. De fait, force est de le constater, notre pays n'a pas les moyens de mettre autant d'argent sur la table que nous le souhaiterions. Après la crise de 2008, vos prédécesseurs, faisant face à une augmentation de la dette, se sont attachés à diminuer le déficit de nos comptes publics. La bien meilleure croissance que vous avez trouvée à votre arrivée pouvait enfin permettre de baisser significativement le niveau de la dette en pourcentage du PIB. Vous vous y étiez d'ailleurs engagés. Malheureusement, à l'orée de cette crise sanitaire, le niveau de la dette était au plus haut ; vous n'en êtes évidemment pas seuls fautifs, mais nous en payons collectivement le prix aujourd'hui. Encore faut-il noter que la politique monétaire plus qu'accommodante de la Banque centrale européenne nous permet, malgré tout, de mener l'action publique nécessaire au moment que nous vivons. J'en viens maintenant à un point qui, pour le groupe socialiste et républicain, est fondamental. Nous nous sommes d'ailleurs régulièrement exprimés sur ce sujet. Au-delà de son coût, c'est la question du paiement de la crise qui nous intéresse. La problématique est d'ailleurs double. En premier lieu - je reviens sur les dépenses sociales -, nous estimons que ce n'est pas au budget social que devrait revenir le paiement des 8 milliards de dépenses de santé liées au Covid-19. Si vous avez, à juste titre, créé une mission budgétaire spécifique dans le budget général, nous estimons que ces sommes devraient y être portées,

Depuis votre arrivée aux affaires, on creuse de nouveau le déficit de la sécurité sociale. Ces dépenses ne sont pas contestables en soi, mais demain, au lieu de faire porter les efforts sur la solidarité nationale, on déremboursera d'un côté, on coupera dans les dépenses de l'autre. de course, ce seront une nouvelle fois les plus précaires, les malades, et nos aînés qui paieront. C'est la raison pour laquelle nous demandons l'inscription de ces dépenses sociales au budget général : la santé d'aujourd'hui ne doit pas se traduire par un affaiblissement de la santé de demain. De plus, s'il devait y avoir une prise en charge par le budget général, nous proposons que, sur le modèle des OPEX, cela se fasse non pas dans l'opacité des décrets de reventilation intraprogramme des crédits, mais, pour partie, dans le cadre d'une solidarité de toutes les missions budgétaires.

Une nouvelle fois, comme après le premier PLFR, nous n'en trouvons guère trace dans votre texte, monsieur le ministre. Lors de l'examen du premier PLFR, vous aviez estimé que ce n'était pas le débat et, malgré nos doutes, nous n'avions pas insisté et avions accepté que le sujet soit renvoyé à plus tard. Nous considérons que plus tard c'est aujourd'hui, et que nous pouvons et devons désormais évoquer les conséquences de cette crise tant pour les finances publiques que pour les particuliers. Le Gouvernement a d'ailleurs déjà ouvert le sujet.

On cherche vainement le « en même temps » cher à notre président. Curieusement, rien sur la solidarité nationale nécessaire, rien sur la participation et l'effort des entreprises, une fois l'activité redémarrée, rien sur la participation des plus fortunés d'entre nous, rien sur la contribution du capital à la restauration de nos comptes. Nous ne repartirons pas avec les recettes du passé ! Nous appelons à davantage de solidarité entre tous et demandons un mécanisme de taxation exceptionnelle du capital. Enfin, on va faire de la politique Une taxation des revenus ou de la consommation serait bien évidemment contre-productive, nous en convenons sans aucune difficulté, eu égard à la spécificité de la crise économique que nous traversons. Cependant, rien sur le plan économique n'empêche la mise en oeuvre d'un mécanisme de solidarité centré sur le capital. Nous vous ferons plusieurs propositions en ce sens durant les débats. Nous n'en doutons pas ! Je sens qu'il y aura des accords Nous nous permettrons également de mettre en lumière certains secteurs d'activité et certaines situations sociales pour lesquelles nous estimons que la réponse du Gouvernement gagnerait à être complétée. En conclusion, monsieur le ministre, nous prenons acte des apports du Gouvernement dans ce deuxième PLFR, notamment pour maintenir le potentiel de croissance de notre économie et faire en sorte sorte que les salariés puissent continuer à vivre et être présents pour la relance. La réponse n'est évidemment pas parfaite, mais elle existe, et le texte gagne en crédibilité par rapport à la première mouture.

d'un blanc-seing, et nous demandons au Gouvernement, dans le cadre de cette lecture au Sénat, d'améliorer sa copie, pour permettre plus de transparence dans la communication et plus de solidarité dans les faits. Messieurs les ministres, je le dis avec gravité, ne prenez pas le risque d'une fracture citoyenne et sociale au lendemain de la crise.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, il y a à peine plus d'un mois, le Sénat adoptait à la quasi-unanimité, rappelons-le, le premier PLFR, dont les dispositions visaient à limiter les effets d'une crise économique sans précédent par son origine

À crise exceptionnelle, moyens exceptionnels ! Il fallait effectivement préserver notre tissu économique et l'emploi, pour préserver notre potentiel de croissance et permettre, le moment venu, un redémarrage le plus rapide possible. Il fallait également éviter qu'une crise sociale ne s'ajoute à la crise sanitaire. Nous avons donc évidemment approuvé ces mesures. Cependant, le vote favorable du groupe Les Républicains ne l'avait pas empêché de formuler plusieurs remarques. les ministres, vos prévisions macroéconomiques nous semblaient alors bien trop optimistes, avec une croissance affichée en recul de 1 % seulement. Les critères d'accès au fonds de soutien aux entreprises nous paraissaient trop restrictifs et présentaient des « trous dans la raquette ». Par ailleurs, le montant de ces aides était faible.

Il manquait également la possibilité de faire un geste de reconnaissance sonnant et trébuchant envers toutes celles et tous ceux qui, par leur engagement à leur poste de travail

la possibilité de primes. Tout cela est bienvenu, monsieur le ministre, et nous l'approuverons, même si notre groupe va proposer un certain nombre d'amendements sur lesquels reviendra Jérôme Bascher. Pour ma part, j'en évoquerai seulement un. Il concerne une question importante, dont vous repoussez encore le traitement : il s'agit de ces milliers d'entreprises qui ne pourront faire face à la crise, même avec les nouvelles dispositions que nous allons adopter. Les plus grandes entreprises, les plus stratégiques, pourront bénéficier du fonds de 20 milliards d'euros que vous créez pour des prises de participations de l'État, voire pour des nationalisations. des autres ? Je pense bien évidemment aux entreprises des secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie et de la culture, dont la reprise d'activité sera encore décalée dans le temps, probablement de plusieurs mois, et pour lesquelles le chiffre d'affaires qui sera perdu le sera définitivement, parce qu'il n'est pas possible de rattraper une saison ratée. messieurs les ministres, et vite. Vous dites être bien conscients du problème, mais vous repoussez la prise de décision. Pourtant, ces entreprises, peut-être plus que les autres, ont besoin d'un minimum de visibilité, parce qu'elles sont les plus fragiles et que leur existence même est en jeu. En ce moment, permettez-moi d'avoir une pensée pour ces artisans, ces commerçants, ces agriculteurs, ces libéraux, ces chefs d'entreprises petites ou moyennes, qui, du jour au lendemain, voient la pérennité de leur activité fortement menacée. Très souvent, c'est l'investissement humain et financier d'une vie. chefs d'entreprise, contrairement à ce que laissent parfois entendre certains, n'est pas un long fleuve tranquille, au bout duquel il n'y aurait qu'à engranger des bénéfices. Eux aussi, du jour au lendemain, ils peuvent tout perdre sans avoir commis la moindre faute de gestion ou la moindre erreur, uniquement victimes des circonstances. Nous devons mesurer

Limiter à 8 % la chute de la croissance, ce que nous espérons tous, dépendra de nombreux facteurs endogènes et exogènes, que vous ne maîtrisez pas tous, messieurs les ministres, ce dont personne ne vous fera le reproche. Si nous voulons avoir une chance de ne pas devoir encore réviser ce chiffre à la baisse, il nous faut très rapidement mettre en place le plan de relance annoncé.

mais le temps n'est pas venu -, pourquoi nous avons tant manqué de masques et de tests, alors que d'autres pays ont pu mettre en place des stratégies différentes et, finalement, limiter bien mieux que nous les dégâts humains et, probablement, économiques de cette crise sanitaire. Sur la base de vos prévisions nouvelles, le déficit public serait donc de 9 % cette année, et le déficit budgétaire d'un peu plus de 186 milliards d'euros après le vote de l'Assemblée nationale. C'est un chiffre considérable, mais c'est le prix que nous devons payer, au risque d'aggraver la crise si nous ne le faisions pas. Cependant, il faut dès à présent penser à l'après. Depuis la crise de 2009, nous n'avons pas su, contrairement à d'autres, inverser la courbe de notre dette en réduisant suffisamment notre déficit public- sans même parler d'un retour à l'équilibre, ce que certains ont fait. Nous avons ainsi perdu dix ans.

Quant à l'Europe, si elle a pris des décisions importantes, chacun voit bien où sont ses limites : les pays du Nord, l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres ne sont pas prêts à accepter l'idée même d'une mutualisation d'une partie de nos dettes. Par ailleurs, l'écart se creuse encore entre nos économies, alors que nous partageons la même monnaie. Il y a là un risque majeur. y a là un risque majeur. Si nous approuvons les mesures que vous prenez pour faire face à cette crise, nous voulons en même temps, dès aujourd'hui, réaffirmer ici que le nouveau « nouveau monde » que le Président de la République nous a annoncé ne pourra pas mettre de côté la question de la dette et du déficit public.

Le dimanche suivant, le Premier ministre annonçait un déconfinement le 11, mais ... Au-delà du jeu de mots, la sortie de confinement est complexe, sans vérité, mais essentielle. Elle doit être précise, car, je le dis solennellement ici, la France ne peut pas se permettre un reconfinement. La reprise en V attendue, un V qui ressemble plutôt au symbole de Nike au fil du confinement, ne ne doit pas être en W puis en L, comme disent les économistes : ce ne serait alors plus une récession, mais une dépression, avec le risque démocratique de sinistre mémoire qui ne manque pas de s'ensuivre. Ce PLFR 2, plus réaliste que la réaction rapide et bienvenue du PLFR 1, Philippe Dallier l'a dit, ne donnera sa pleine efficacité que sous deux conditions, déjà évoquées dans le de Descartes. Pour réussir le déconfinement, il faut donner de la clarté et un calendrier, secteur par secteur, mais aussi pays par pays, car, vous l'avez dit, monsieur le ministre, tout doit être coordonné. J'ai peur que l'Union européenne ne passe à côté de l'histoire. L'incertitude et les palinodies sont les armes létales de la reprise. Donnons vite des perspectives avec un PLFR 3, véritable pacte de stabilité et de croissance il convient d'écouter et de réagir aux manques que ce plan globalement bien construit et bien calibré laisse entrevoir, malgré votre bonne volonté. J'en viens à l'esprit qui nous anime remonter les inquiétudes de l'économie réelle oubliées par les administrations centrales, les fameux « trous dans la raquette » des aides. La commission des affaires économiques, sous l'impulsion de Sophie Primas, comme celle des finances, avec Vincent Éblé et Albéric de Montgolfier, mais aussi celle des

Car c'est notre grande conviction : les efforts de crise doivent être partagés par tous, banquiers et assureurs, grandes surfaces, État et collectivités, mais aussi contribuables et travailleurs de tout type, syndicats, qui doivent jouer le jeu du travail et du dialogue.

raccourcir les délais pour engager plus vite les chantiers, relever le plafond de défiscalisation des dons et du mécénat liés à la crise sanitaire, baisser la TVA sur les masques et les gels hydroalcooliques, ... C'est fait ! ... surtout lorsque ce sont les collectivités qui les financent à la place de l'État.

des prises de participation, je crois plus à celles de Bpifrance et de la Caisse des dépôts et consignations qu'à celles de l'État, qui se révèle souvent un bien mauvais actionnaire,

Il s'agit tout d'abord du calendrier et des perspectives économiques dans les semaines et les mois à venir. Je souhaite que nous puissions procéder étape par étape, ne serait-ce que par souci de clarté vis-à-vis des Français. Le premier temps a été celui de la riposte économique : c'est le plan d'urgence économique que nous avons mis en place et qui est amélioré par ce projet de loi de finances rectificative, lequel tient compte, je le répète, des remontées du terrain, des critiques, des observations et des propositions.

pratiques, sous quelles conditions pourront se rouvrir un certain nombre de commerces. Ce deuxième temps s'étalera sur plusieurs semaines. Il durera un peu plus longtemps pour certains secteurs comme la restauration, qui sont soumis, nous l'avons tous dit, à des contraintes particulières. Le troisième temps sera celui de la relance économique. À mon avis, rien ne serait pire que de mélanger les différentes étapes, ne serait-ce que vis-à-vis de nos compatriotes. La riposte est immédiate la reprise aura lieu dans quelques jours pour un certain nombre de secteurs économiques ; et la relance est située à un horizon de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, pour être efficace, bien calibrée et coordonnée avec nos partenaires européens.

n'a jamais été notre position. Vous pouvez reprendre toutes mes déclarations depuis plusieurs semaines, j'ai toujours indiqué que la reprise économique serait lente, longue et coûteuse, et je ne retire pas un seul de ces mots. mots. Selon moi, le discours de vérité est le bon discours vis-à-vis des Français. C'est vrai, cette crise est sans précédent dans notre histoire économique récente. Dans son intensité, elle n'est comparable qu'à la grande récession de 1929. 1929. Retrouver des niveaux de croissance économique et de prospérité comparables à ceux que nous avons connus prendra du temps, sera difficile et coûteux. Il vaut mieux le dire dès le départ. Les raisons en sont très simples et très pratiques.

Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le cobalt, qui permet de fabriquer des batteries électriques ! La République démocratique du Congo a confiné un certain nombre de ses mines dans lesquelles est extrait le cobalt. Ainsi l'approvisionnement en matières premières va-t-il s'avérer compliqué.

Enfin, troisième raison, la reprise sera lente, difficile et coûteuse parce qu'elle devra s'accompagner de règles sanitaires strictes.

un langage de vérité. La discussion générale est close. Mes chers collègues, compte tenu du nombre d'amendements déposés, à savoir 339, et afin d'organiser nos travaux dans de bonnes conditions, je vous propose de suspendre la séance jusqu'à Monsieur le président de la commission des finances, pouvez-vous nous indiquer l'heure à laquelle vous souhaitez réunir la commission ? Je propose que la commission se réunisse à dix-neuf heures. Il y a en effet un délai nécessaire à l'élaboration du dérouleur par les services de la séance.